La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du mardi 31 juillet

Je tiens également à saluer notre nouveau collègue Damien Regnard, qui est devenu sénateur le 28 juillet dernier. L'ordre

le navire humanitaire a demandé hier à la France, « à titre exceptionnel », de pouvoir débarquer à Marseille les 58 migrants secourus à son bord, dont 18 enfants. Les autorités maritimes panaméennes ont annoncé samedi qu'elles allaient retirer son pavillon à l', déjà privé de pavillon par Gibraltar, l'État de Panama indiquant que la principale plainte émanait des autorités italiennes. Les ONG SOS Méditerranée et Médecins sans frontières ont dénoncé « la pression » exercée par le gouvernement italien sur le Panama. Dans ce contexte, le ministre Bruno Le Maire, interrogé ce matin, a rappelé la « position de fermeté du Gouvernement ». Très préoccupé par ce sujet, le groupe socialiste et républicain demande qu'un débat sur la politique de la France au regard de cette urgence humanitaire soit inscrit à l'ordre du jour du Sénat. Mais, dans l'immédiat, nos questions sont les suivantes. Depuis 2014, des milliers de migrants trouvent la mort chaque année en Méditerranée, et désormais l'Italie et Malte ont décidé de fermer leurs ports. Quelle va être la réponse définitive du Gouvernement à la demande de l'de débarquer à Marseille ces 58 naufragés ? Quelle est, également, l'appréciation du Gouvernement de la demande italienne faite au Panama de retirer le pavillon au dernier bateau humanitaire assurant des sauvetages en Méditerranée ? Face à cette pression, qui s'exerce à l'encontre des ONG et de leurs actions, n'est-ce pas une façon de se défausser que d'attendre qu'une « solution soit trouvée au niveau européen », pour reprendre les éléments de langage diffusés largement par plusieurs ministres ce matin ? La parole

le navire a recueilli, au total, 58 migrants en mer, au large des côtes libyennes. Ces interventions de l'ont menées en devançant les garde-côtes libyens, qui se dirigeaient eux aussi vers les embarcations signalées, pour leur porter secours. La nuit dernière, l's'est une nouvelle fois dirigé vers une embarcation transportant 120 migrants, alors même que les garde-côtes libyens ont finalement pu leur porter assistance. L's'est désormais éloigné des côtes libyennes et est à la recherche d'un port de débarquement. Or, comme vous l'avez dit, nous apprenons que le Panama lui a retiré son pavillon. Le navire se situe actuellement à 100 milles nautiques au sud de l'île de Malte. Il entre dans la zone de sauvetage sous la responsabilité de Malte. le droit de la mer prescrit que les navires ayant recueilli des naufragés en mer doivent les débarquer dans le port sûr le plus proche. L'doit respecter cette exigence, afin d'épargner aux hommes, aux femmes et aux enfants présents à bord que la navigation se prolonge inutilement. Il va de soi

Comme nous le faisons chaque fois, nous ferons notre devoir

et Territoires. Monsieur le ministre de l'intérieur, depuis quelques semaines bruissent des rumeurs sur un projet d'absorption des compétences départementales par les métropoles. Comme je me méfie des rumeurs, qui sont souvent irréversibles et incontrôlables, je préfère m'adresser directement à vous pour connaître leur bien-fondé. Ce ne serait pas la première fois qu'un gouvernement ambitionne une grande réforme territoriale. des plans de décentralisation, de la volonté de fusionner département et région. Nous gardons en mémoire le territorial de Manuel Valls. Quel succès ça a été ! Chaque gouvernement a sa nouvelle géographie de la France. Lors de sa campagne électorale, l'actuel Président de la République a inscrit dans son programme l'idée de supprimer les départements dont les compétences seraient transférées aux métropoles. en s'inspirant des districts métropolitains du Royaume-Uni, de concentrer les efforts autour de quelques pôles, sortes de locomotives dont la vocation serait de tirer les territoires vers le haut. Mais qu'est-ce qui nous garantit que les wagons suivront Quels sont les rouages qui permettront aux territoires les plus reculés de bénéficier du rayonnement économique, social, culturel de ces nouvelles mégapoles ? Le Grand Lyon a avalé, depuis 2015, les compétences du département du Rhône. Aujourd'hui seraient concernés les villes de Lille, Nantes, Nice, Toulouse et Bordeaux et, donc, les départements du Nord, de Loire-Atlantique, des Alpes-Maritimes, de Haute-Garonne et de Gironde. Sans préjuger du bien-fondé de cette réflexion et de l'opportunité d'une réforme, l'ancien conseiller général que je suis formule trois interrogations fondamentales quelle représentativité accorderiez-vous aux zones rurales ? Pensez-vous que les métropoles aient la culture sociale chère aux départements ? Quel serait le mode opératoire ?

part, je ne suis pas de ceux qui opposent les zones rurales et les zones métropolitaines. Je pense qu'il y a la place pour les unes et pour les autres.

tandis que d'autres sont centrées sur elles-mêmes. C'est cela, le véritable problème ! Il faut donc construire des partenariats entre les métropoles et l'ensemble des territoires qui les environnent. C'est cela, l'ambition du Gouvernement

Le week-end dernier, le centre-ville d'Angers a été saccagé ; les forces de l'ordre ont été prises en étau, si je puis dire, à La Roche-sur-Yon ; 26 % des femmes n'osent plus sortir, par crainte d'une agression- c'est l'Observatoire national de la délinquance qui le dit. Pendant ce temps-là, nos forces de l'ordre manquent cruellement de moyens. Des gendarmes me disaient récemment qu'ils n'ont même plus de gazole à mettre dans leur véhicule pour effectuer leurs sorties quotidiennes. ... Quand allez-vous donner enfin des moyens à nos forces de l'ordre ? Je suis même tenté de vous demander : comment allez-vous faire pour reprendre en main une situation qui semble cruellement vous échapper ?

le Président de la République avait annoncé, pendant sa campagne électorale, que nous allions, durant ce quinquennat, créer 10 000 postes dans la police et la gendarmerie,

de budget pour 2019 s'inscrit dans la même ligne : dans un contexte financier que vous savez difficile, le budget des forces de sécurité intérieure atteindra 13,1 milliards d'euros, en augmentation

une seule obsession : la sécurité des Français. C'est comme ça qu'on réussit ! C'est place Beauvau qu'on donne l'exemple ! La sécurité, c'est une question de moral. Aujourd'hui, le moral des troupes n'y est pas, parce qu'elles attendent un chef qui soit à leur disposition vingt-quatre heures sur vingt-quatre et qui n'ait pas la tête ailleurs

Pourtant, ces soldats du feu, ces hommes et ces femmes dont le courage et le dévouement sont exemplaires, n'ont pas choisi de s'engager au service de nos concitoyens pour être pris pour cibles, menacés ou agressés. La menace qui pèse sur nos sapeurs-pompiers ne se limite pas à l'atteinte à leur intégrité physique : leur statut pourrait également être remis en cause. En effet, nos sapeurs-pompiers volontaires sont visés par une directive européenne portant sur le temps de travail, dont la transposition en droit français remettrait en cause le volontariat comme engagement altruiste et généreux. Dans ce contexte, l'efficacité de notre modèle de sécurité civile serait profondément réduite, ce qui condamnerait irrémédiablement le travail réalisé dans le cadre de la mission volontariat, à laquelle notre collègue Catherine Troendlé a participé en tant que rapporteur. Monsieur le ministre d'État, une initiative forte auprès des instances de l'Union européenne semble urgente et indispensable pour exempter le volontariat de cette directive, ou éventuellement obtenir des dérogations adaptées. Faut-il rappeler que le Président de la République avait pris l'engagement « de défendre farouchement le modèle reposant sur le volontariat des sapeurs-pompiers, qui n'est ni du salariat ni du bénévolat »

Le Sénat s'est mobilisé fortement en cosignant très majoritairement une motion qui sera adressée prochainement à Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne. européenne. Ainsi, à la veille du congrès national des sapeurs-pompiers de France, quelles mesures ou initiatives concrètes entendez-vous prendre pour préserver notre modèle de sécurité civile, le volontariat, et assurer la protection de nos sapeurs-pompiers et de nos concitoyens ?

Ce phénomène de sécheresse, qui a débuté en juin, touche particulièrement les éleveurs. Il a fallu nourrir le bétail dans les prés dès le mois de juillet, et les stocks de fourrage, alors qu'ils sont destinés à l'hiver, sont déjà bien entamés 20 % à 40 % des prairies naturelles, qui sont autant de réservoirs à fourrage, ont été brûlées par le soleil. Pour ce qui concerne les cultures de soja et de maïs, le manque d'eau a engendré jusqu'à 40 % de perte de rendement. Pour de nombreux exploitants agricoles, le colza a été incapable de lever faute d'une pluviométrie suffisante. Éleveurs et agriculteurs, aux quatre coins du pays, se trouvent aujourd'hui dans une situation intenable. Afin d'éviter une catastrophe économique dans les territoires ruraux, il est urgent que l'État mette en oeuvre des dispositifs pour les aider, sans faire porter la solidarité uniquement par l'Europe ou par les agriculteurs eux-mêmes. M. le ministre de l'agriculture a déjà annoncé que des avances sur la PAC seront touchées dès la mi-octobre, à hauteur de 70 % sur le premier pilier et de 80 % sur le second pilier. Il a également annoncé un dégrèvement de la taxe sur le foncier non bâti et un report des paiements des cotisations sociales auprès des caisses de la MSA,

Les services de l'État ont anticipé cette situation. Dès le mois de juillet, Stéphane Travert a annoncé la mise en oeuvre de mesures nationales activables dans tous les départements, de façon individualisée selon l'aléa climatique : exonération de la taxe additionnelle sur le foncier non bâti sur les parcelles touchées,

Des autorisations telles que la possibilité de faire pâturer ou faucher les surfaces en jachère ont également été accordées. Les autres aides de soutien en cas d'aléas climatiques seront versées au fur et à mesure de la reconnaissance des situations individuelles. Madame la sénatrice, sachez que Stéphane Travert a donné des instructions précises aux préfets, afin d'établir un état des lieux département par département. Ce retour aura lieu dans quelques jours, début octobre. Bien entendu, il faudra que le Gouvernement reste, comme il l'a été jusqu'à présent, totalement mobilisé

L'une des mesures essentielles du projet de loi de finances pour 2019, c'est une meilleure rémunération du travail par la baisse des charges. J'approuve ces orientations, mais je suis au regret de constater que le budget du ministère de l'agriculture fait tout le contraire. En supprimant l'exonération des charges patronales sur les emplois saisonniers, on signe la fin de l'agriculture, en particulier de la petite agriculture

La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances. Monsieur le sénateur

Dans ce contexte, il était logique de remettre à plat les dispositifs spécifiques. C'est pourquoi le régime TODE a été concerné : dans le cadre du renforcement opéré au titre du régime général, ce régime gagne en attractivité, et les dispositifs spécifiques deviennent moins justifiés. L'impact global de la réforme générale est positif en année pleine, avec un gain de 60 millions d'euros nets pour l'agriculture, les coopératives et les industries agroalimentaires françaises. Cet impact global recouvre des réalités différentes : un gain important pour la coopération et la transformation affiliées au régime agricole, mais, dans certains secteurs, en particulier le maraîchage, l'arboriculture et la viticulture, la suppression du dispositif TODE aura- et nous ne l'ignorons pas -des conséquences.

L'analyse d'ensemble doit tenir compte des gains induits par les autres mesures annoncées la semaine dernière : la réforme de la fiscalité agricole ; la mesure relative à l'épargne de précaution, permettant de mieux appréhender la variabilité du revenu des agriculteurs ; l'exemption des agriculteurs de la hausse de la TICPE, la taxe C'est dans le cadre de cette analyse d'ensemble que nous recevrons les représentants des organisations professionnelles, afin d'envisager des mesures spécifiques pour répondre aux inquiétudes qui subsistent.

Notre société est minée par des inégalités croissantes- les rapports successifs de nombreux observateurs le démontrent régulièrement. Du côté de la distribution de dividendes, les groupes français- les plus généreux au monde -ont versé 47 milliards d'euros au deuxième trimestre de cette année. Sur 100 euros de bénéfices, 67 vont aux actionnaires, 5 seulement aux salariés avez annoncé hier vouloir redistribuer du pouvoir d'achat aux salariés et retraités de ce pays, mais, dans le même temps, vous annoncez 4 100 suppressions de postes de fonctionnaires, dont 1 800 dans la seule éducation nationale. En matière d'éducation, on ne dépense pas : on investit pour l'avenir et pour la productivité ! Quant aux 2 227 suppressions de postes annoncées dans l'administration fiscale, ce seront autant de moyens de contrôle en moins pour lutter efficacement contre l'évasion fiscale. M. le ministre de l'économie a dit hier en commission : on ne peut pas distribuer la richesse que l'on n'a pas. Le constat est fait que la richesse, nous l'avons. Ce qui manque, c'est la redistribution Gel du point d'indice des fonctionnaires, hausse des retraites bloquée à 0,3 %, qui entraînera d'office une baisse du pouvoir d'achat, déjà amputé cette année par la hausse de la CSG, et hausse des prix du tabac et du carburant- cette liste n'est pas exhaustive. Redonner du pouvoir d'achat passe d'abord par une augmentation sensible du SMIC, une revalorisation des pensions et une mise à contribution des dividendes en croissance forte. La suppression de l'ISF et la création de la à 30 % n'ont, à l'évidence, pas permis de s'attaquer frontalement aux inégalités. La théorie du ruissellement, à laquelle vous semblez croire encore, n'a jamais fait, nulle part, la preuve de son efficacité : Anne, ma soeur Anne, ne vois-tu rien venir ? Mesdames, messieurs les ministres, quand allez-vous enfin tourner le dos aux politiques d'austérité ? La parole est à M. le Premier ministre.

que nous fixons pour l'action de l'État et les défis que nous devons relever. Le premier bloc à connaître une augmentation réelle des moyens qui lui sont affectés est celui qui concerne la sécurité des Français. La défense nationale,

de sécurité publique, de protection contre le terrorisme et d'amélioration de notre système judiciaire sont au coeur de notre pacte républicain. Je crois, monsieur le sénateur, que, sur ce point, vous êtes d'accord avec nous. Le deuxième grand bloc de mesures qui vont voir leurs moyens augmenter, ce sont les investissements pour l'avenir.

en matière de politique du logement, la décision que nous avons prise de passer à la juste prestation, c'est-à-dire à la « contemporanéisation » du versement des APL, nous permettra

à ce qu'on appelle la « sincérisation », à laquelle la Cour des comptes nous avait vivement encouragés, après, peut-être, des relâchements trop prononcés dans le passé- remarquez que je le dis avec mesure.

champion du monde de la communication dans beaucoup de domaines ! Eh oui ! Pour le sport, vous ambitionnez quatre-vingts médailles pour 2024, trois millions de nouveaux pratiquants, une nouvelle gouvernance et un budget préservé. Nous partageons ces ambitions, mais nous faisons face aussi à vos contradictions : le budget des sports représente moins de 0,2 % du budget national et diminue fortement, 451 millions d'euros en 2019. Sans oublier la suppression de la réserve parlementaire, qui finançait nombre de manifestations et équipements sportifs sur notre territoire. est aujourd'hui la triste réalité de votre politique sportive ! Madame la ministre, vous avez demandé au mouvement sportif de vous faire confiance, mais, face à vos annonces, ce sont désormais des milliers de bénévoles et de clubs, soutenus, je le rappelle, à hauteur de 12 milliards d'euros par an par les collectivités territoriales, qui se retrouvent dans l'incertitude. Les solutions existent ; le Sénat les a déjà proposées voilà un an. Il s'agit que le sport finance le sport et que les taxes affectées soient enfin déplafonnées, contrairement aux choix que vous nous proposez.

accepterez-vous de déplafonner les taxes sur les jeux et la taxe Buffet, afin que le budget des sports retrouve son niveau de 2017 ?

Monsieur le sénateur Savin, je vous remercie de votre question et de l'intérêt que vous portez au budget du ministère des sports. Je vous rejoins sur un point : les enjeux de la politique sportive sont nombreux. Je porte, moi aussi, cette ambition, tant pour le rayonnement du haut niveau que pour l'accès aux pratiques sportives pour tous les publics et sur tout le territoire.

nous conserverons les mêmes moyens d'intervention qu'en 2018, une capacité d'action intacte et la même volonté d'agir en faveur du sport français. Monsieur Savin, vous savez, j'en suis sûre, que, dans le budget pour 2018, le poste relatif à la compensation de l'exonération des cotisations salariales des arbitres a été surévalué de 40 millions Dans le projet de loi de finances, dont la première caractéristique, que vient de rappeler M. le Premier ministre, est d'être sincère, 30 millions d'euros apparaissent en effet en différentiel, et je l'assume.

notamment du lissage des dépenses sur les grands événements sportifs et de la fin des programmes d'investissement, par exemple pour la restructuration de l'INSEP. Cette enveloppe globale de 40 millions d'euros- 10 d'une part, vers la haute performance et, d'autre part et surtout, vers le développement des pratiques : 25 millions d'euros pour la haute performance et 15 millions d'euros supplémentaires alloués à la réduction des inégalités d'accès à la pratique sportive sur les territoires carencés, notamment à travers le renforcement du savoir nager, un sujet qui, vous le savez, me tient à coeur. À ce propos, mesdames, messieurs les sénateurs, j'attire votre attention sur le fait que nous poursuivons les discussions afin d'obtenir des financements supplémentaires pour réduire encore les inégalités territoriales.

votre budget baisse de 30 millions d'euros. Une nouvelle fois, ce sont les arbitrages de Bercy qui ont eu gain de cause, et non le budget du sport. Eh oui ! Le Sénat fera donc son travail, en réaffectant les crédits nécessaires pour qu'une politique sportive sur l'ensemble des territoires puisse perdurer : c'est ce qu'attendent le milieu sportif et l'ensemble de ses bénévoles !

écologique et solidaire. Le 25 septembre 2015, voilà trois ans, 193 États membres adoptaient à l'ONU le programme de développement durable à l'horizon de 2030, dit Agenda 2030. Cet agenda est porteur d'une vision forte : transformer le monde en affichant l'éradication de la pauvreté comme une nécessité et se donner les moyens d'une transition vers un développement durable. Dix-sept objectifs de développement durable et 169 cibles ou sous-objectifs forment le coeur de cet agenda, qui engage ses signataires. Une partie de ces engagements Sur ce sujet, la France est en première ligne. Le 24 novembre dernier, à l'occasion du congrès des maires, le Président de la République annonçait le lancement des assises de l'eau, afin notamment de renouveler et de moderniser nos infrastructures. En avril dernier s'ouvrait la première séquence de ces assises, consacrée à la relance des investissements sur les réseaux et l'assainissement. Dans ce cadre, et pour répondre au mieux aux attentes des territoires, une concertation très large et inédite a été engagée avec les élus locaux, notamment une consultation en ligne des maires et des échanges sur le terrain au sein des comités de bassin. Cette méthode était claire : s'appuyer sur les élus locaux pour être au plus proche des préoccupations de nos concitoyens. En parallèle, un diagnostic détaillé révélait notamment qu'un litre sur cinq se perd dans les réseaux d'eau, avec de forts contrastes selon les services d'eau et d'assainissement. Il ressort des assises de l'eau que, pour améliorer la qualité de service et optimiser les investissements, il faut améliorer la connaissance des services d'eau sur l'ensemble du territoire. En définitive, ces assises de l'eau, en s'appuyant particulièrement sur les élus locaux, ont été riches d'enseignements.

et un investissement inédit, sur lequel le Premier ministre lui-même a présenté des annonces dans les Hautes-Alpes, au début de ce mois. Le premier principe, c'est l'attachement collectif au principe et au modèle des agences de l'eau, avec à leur côté leur conseil d'administration et les différents comités de bassin. Le deuxième principe, c'est l'affirmation des solidarités

Pendant dix ans, j'ai exercé le beau mandat de maire dans une petite commune de montagne. Très présente sur le terrain, je constate la résignation qui gagne les maires et, plus largement, l'ensemble des élus municipaux. Baisse des dotations, suppression de la taxe d'habitation, diminution des contrats aidés, changements incessants des lois et réglementations, inflation des normes techniques coûteuses, fermeture des services publics, irrespect des lois et violences par les gens du voyage : la liste est longue des problèmes qui expliquent le ras-le-bol des maires. Des maires qui souffrent de ne pas se sentir considérés par l'État, dont ils sont pourtant les premiers serviteurs. Des maires qui, eux, établissent et font voter des budgets en équilibre, quand l'État, lui, n'a pas présenté un budget en équilibre depuis 1974. Des maires qui en ont assez d'être pointés du doigt par l'État pour leur gestion, alors qu'ils gèrent leur commune en bons pères de famille. Cet été, un chiffre est passé inaperçu : plus de 1 000 démissions de maires ont été recensées depuis 2014. Gageons que, en 2020, malheureusement, ils seront nombreux à ne pas se représenter. Aujourd'hui, monsieur le ministre d'État, les maires se posent des questions sur l'avenir du mandat municipal, et nous avec eux. Quand un député parisien de votre majorité déclare cet été qu'il suffit de regrouper les communes, que cherche-t-on : une République de « technotables Demain, comment le Gouvernement pourra-t-il réformer le pays sans le concours des communes et de leurs élus, alors que l'État n'a plus assez de services sur le terrain ? Comme le répète inlassablement le président du Sénat, l'État ne peut se réformer contre les territoires Notre République a besoin des communes, qui constituent le terreau de la démocratie. Les maires en sont les vigiles autant que les fantassins. Monsieur le ministre d'État, ma question est simple : le Gouvernement est-il prêt à changer d'attitude et de cap pour renouer le dialogue avec les maires de France et leur redonner leur place, leur rôle et leurs moyens d'action légitimes au service du pays ?

Madame la sénatrice, permettez-moi de vous féliciter pour votre élection au Sénat de la République. de la République. Je connais bien votre département, pour y être allée régulièrement. J'ai de nombreux amis élus en Haute-Savoie, et j'y pensais en écoutant la réponse précédente, car j'étais tout à fait dans votre secteur au mois de mars,

travailler avec les élus locaux et construire des politiques avec eux. C'est en effet dans le dialogue, madame la sénatrice, que le Gouvernement agit sur le terrain et négocie au sein de la Conférence nationale des territoires,

La parole est à M. Vincent Éblé, pour le groupe socialiste et républicain.

puis devant les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le travail des semaines à venir sera utile pour lever les interrogations qu'un document aussi déterminant ne manquera pas de susciter chez bon nombre d'entre nous et chez nos concitoyens. Il est de tradition de faire porter la communication gouvernementale sur quelques mesures phares, mais le parlementaire expérimenté s'efforcera de reconstituer par consolidation la réalité des grands équilibres et de gommer les effets de périmètre et de transferts, importants cette année, en particulier

-et réformes nouvelles propres à l'année 2019. À l'évidence, les analyses convergent : sauf pour les catégories sociales à fort revenu, la note sera salée Je pense aux familles, aux ménages, aux consommateurs. Je pense, bien entendu, aux retraités : avec la hausse de la CSG combinée au rabot sur les retraites, 4,5 millions de retraités sur les 7 millions qui ont subi cette hausse resteront perdants en 2019. Je pense aussi aux ruraux et périurbains confrontés pour leurs déplacements à une hausse soutenue de la fiscalité énergétique et indirecte, qui pèsera sur leur pouvoir d'achat l'an prochain Madame la secrétaire d'État, dans une période où notre croissance économique reste supérieure à la croissance potentielle, des marges de manoeuvre existent que nous n'avions pas par le passé : n'est-ce pas l'occasion de mener une politique fiscale plus juste entre les Français ?

dont les hypothèses ont été reconnues comme vraisemblables et crédibles par le Haut Conseil des finances publiques et qui a été construit sur des bases clarifiées en 2018. C'est aussi un budget fidèle à notre cap, à nos engagements et à nos priorités. Il nous permet de tenir nos engagements européens en matière de finances publiques, avec un déficit pour la troisième année consécutive en dessous des 3 % du PIB, et de tenir les engagements du Gouvernement en matière de trajectoire pluriannuelle, avec des allégements d'impôts et de prélèvements significatifs, en particulier sur les ménages, qui bénéficieront d'un allégement de prélèvements de 6 milliards d'euros

comme vous avez insisté sur ce point, qu'il permet aussi de protéger les plus modestes et les plus vulnérables, qui bénéficieront de la suppression de la deuxième tranche de la taxe d'habitation, ainsi que de la revalorisation du minimum vieillesse

Sur ces éléments, je pense, monsieur le président Éblé, que nous aurons une discussion équilibrée en commission. La parole est à M. Vincent Éblé, pour la réplique. Madame la secrétaire d'État, vous pouvez tenter de masquer la réalité en rendant les évidences invisibles, mais les contribuables français modestes savent compter ils ne sont pas dupes des jeux de bonneteau où l'on reprend d'une main le double de ce que l'on a donné de l'autre

La séance est reprise. J'ai le regret de vous faire part du décès de nos anciens collègues Josy Moinet, qui fut sénateur de la Charente-Maritime de 1973 à 1989, Robert Vizet, qui fut sénateur de l'Essonne de 1986 à 1995, et Philippe Arnaud, qui fut sénateur de la Charente de 1996 à 2008. Par lettre en date du 19 septembre 2018 et conformément à l'article 22 du règlement, M. Hervé Maurey, président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, a indiqué à M. le président du Sénat que la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable demande au Sénat, en application de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, de lui conférer les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête pour une durée de six mois, afin de mener sa mission d'information sur la sécurité des ponts. Cette demande sera examinée par la conférence des présidents lors de sa réunion de ce soir. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique est parvenue à l'adoption d'un texte commun. J'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de la commission de la culture et de la commission des affaires économiques ont été publiées. Aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 8 du règlement ne s'étant manifestée, ces candidatures ont été ratifiées. J'informe le Sénat que des candidatures ont été publiées pour siéger au sein des commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi et de la proposition de loi organique relatives à la lutte contre la manipulation de l'information.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

dans cette enceinte pour débattre en nouvelle lecture du projet de loi dit « ÉGALIM ». Je le sais, il ne s'agira que d'un simple échange de vues, à la fois sur la méthode, que vous regrettez, et sur le fond du projet de loi que, visiblement, vous jugez insuffisant, inopérant et trop contraignant. Le débat ne se poursuivra donc pas au-delà de la discussion générale.

Notons d'ailleurs que près d'une trentaine d'articles ont été votés conformes par l'Assemblée nationale et le Sénat, soit plus d'un quart des articles du projet de loi. Une soixantaine d'articles restaient encore ouverts à la discussion, mais vous n'avez pas souhaité prolonger les débats.

Les inquiétudes que vous formulez sont de deux natures : il y a d'abord le caractère selon vous inopérant du titre I, destiné à transformer durablement les relations commerciales au sein de la chaîne de production alimentaire ; il y a ensuite les surcoûts et charges induits par le titre II relatif à la qualité de notre alimentation.

qui voudrait des réponses immédiates sur tous les sujets, et, d'autre part, une capacité de transformation de nos modèles agricoles qui doit tenir compte du contexte économique et social. le titre I, votre majorité dénonce un recul, un manque d'ambition. Je ne suis évidemment pas d'accord et n'ai pas changé d'avis. Le projet de loi, je le rappelle, traduit les conclusions des États généraux de l'alimentation, les résultats des ateliers 5 à 7 au sein desquels tous les acteurs présents avaient parfaitement en tête un certain nombre de contraintes juridiques et économiques. Il importe de les garder à l'esprit, y compris au moment de légiférer. Je l'ai déjà indiqué ici même, et nous en avons déjà largement débattu en première lecture : si l'idée est de fixer les prix agricoles ou d'imposer des prix planchers, je le reconnais bien volontiers, le Gouvernement ne le fera pas ! En effet, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes intégrés dans une économie de marché. Si l'idée est de contraindre vendeurs et acheteurs à utiliser tel ou tel indicateur dans la construction des prix, je le dis là encore : le Gouvernement ne s'est pas engagé dans cette voie, car il est le garant du respect du droit national et européen, du droit de la concurrence et de la liberté contractuelle. Alors, de quoi est-il question ? Ce qui se joue en vérité, c'est une transformation en profondeur de la culture contractuelle dans les filières agricoles. Se convaincre de l'intérêt de la contractualisation, de la mise par écrit des engagements réciproques, de l'objectivation des coûts de production et des valorisations de marché, c'est cela le changement de paradigme que je recherche au travers de ce projet de loi ! Il s'agit de s'en convaincre, puis de se donner les moyens d'y parvenir grâce à un cadre juridique nouveau, celui que pose la loi, et un travail de fond entre les différents acteurs économiques. J'ai bien compris que c'est ce travail qui inquiète beaucoup.

lorsqu'on repense la segmentation d'un marché, on se rende parfois compte qu'il manque souvent un ou deux indicateurs pour valoriser un effort de montée en gamme, une production sous label rouge ou bio. Avoir conscience de ce qui existe et de ce qui manque, c'est déjà progresser. Il faut ensuite se fixer une méthode et un calendrier pour combler les lacunes et avancer. Les filières, que j'ai rencontrées durant les semaines passées, se confrontent actuellement à ce questionnement. Elles posent des questions techniques. Elles essaient aussi de construire du consensus entre leurs maillons sur les déterminants économiques de leur fonctionnement : qu'est-ce qui pèse sur les coûts de production de l'éleveur ? Le coût de l'alimentation animale, bien sûr ! Quoi d'autre ? Qu'est-ce qui vient peser sur les prix au stade de l'abattage ? Et aux stades suivants

L'État ne se désintéresse évidemment pas du sujet des indicateurs. Au contraire, le Président de la République a rappelé dès cet été que le volet économique des plans de filière et le projet de loi devaient avancer du même pas. Tout se tient : l'inversion de la contractualisation, qui est dans la loi, le choix des indicateurs, qui incombe aux professionnels, et la régulation de l'aval- l'encadrement des promotions et le seuil de revente à perte -, qui se fera par voie d'ordonnance. Si chacun fait son travail et défend ce projet commun, celui qui faisait consensus pendant les États généraux de l'alimentation, celui d'un rééquilibrage des relations commerciales et d'une meilleure rémunération des maillons les plus faibles de la chaîne alimentaire, je peux vous dire que ce projet ira à son terme Je dis régulièrement, et je veux insister sur ce point encore aujourd'hui, que la loi n'est que l'un des outils de mise en oeuvre de la politique de l'alimentation présentée par le Premier ministre en clôture des États généraux le 21 décembre dernier. Il y en a d'autres, et pas seulement les plans de filière. C'est cet ensemble d'outils que nous devons construire simultanément pour pérenniser et transformer notre agriculture, et enfin répondre aux attentes de nos concitoyens. Jour après jour, nous avançons. Je voudrais vous donner quelques exemples de caps franchis collectivement depuis l'examen du projet de loi en première lecture.

dans le domaine agricole. Le 27 juillet, lors de la réunion du comité d'orientation stratégique Écophyto, a été lancé le plan Écophyto II+, qui contribuera à la réduction de la consommation des produits phytopharmaceutiques. D'autres actions ont été mises en oeuvre. Je pense, par exemple, à la réforme fiscale que nous avons engagée avec Bruno Le Maire en février dernier, à laquelle des parlementaires de toutes les sensibilités ont été associés. Celle-ci permettra d'améliorer

Je pense aussi à l'ingénierie financière pour mettre en place, avec le Fonds européen d'investissement, un fonds de garantie de 800 millions d'euros. Ce fonds permettra de garantir les prêts aux exploitations agricoles,

ma volonté farouche de redonner de la fierté à nos producteurs, un environnement d'action porteur, un cadre juste et équitable à tous les maillons de la chaîne alimentaire. C'est une volonté tout aussi ferme d'assurer à tous nos concitoyens une alimentation toujours plus saine et répondant à leurs attentes légitimes. Promouvoir la performance économique, environnementale, sanitaire et sociale de l'agriculture, comme je le fais à chacun de mes déplacements en France comme à l'étranger, c'est concret. C'est travailler sur la viabilité économique des exploitations, leur résilience, la qualité de l'eau et de l'air, la préservation des sols et de la biodiversité, l'atténuation du changement climatique, la sécurité sanitaire du producteur au consommateur. C'est aussi veiller à ce que les efforts sur la qualité de l'alimentation bénéficient à tous, y compris aux plus modestes de nos concitoyens. Cette quadruple performance s'applique à tous les maillons, dont les industries agroalimentaires.

et de l'accompagnement, celle de la construction de compromis, en impliquant tous les acteurs dans leurs responsabilités. Changer les pratiques peut faire peur, c'est humain. Notre rôle, celui du Gouvernement, mais aussi le vôtre, est de mobiliser, de faire connaître, de diffuser d'autres méthodes pour montrer que la transformation de nos systèmes agricoles vers des modèles plus durables et plus résilients est possible, mais qu'elle ne se fera pas sans ceux qui travaillent la terre

saisissez-vous des outils qu'offre la loi. Elle est un cadre d'action, il vous appartient de l'occuper. Regroupez-vous en organisations de producteurs et en associations d'organisations de producteurs pour être plus forts. Agissez au sein de votre interprofession pour qu'elle élabore et diffuse les indicateurs les plus adaptés à vos filières. Appuyez-vous sur ces indicateurs de référence dans vos propositions de contrat et sur le poids que leur conférera la validation de l'interprofession. C'est comme cela que vous pourrez faire bouger les lignes dans vos relations contractuelles. C'est bien là l'esprit des États généraux de l'alimentation. S'agissant du titre II, ramener du revenu dans les exploitations

Je voudrais m'arrêter quelques instants sur des sujets importants, qui ont été l'objet d'intenses discussions dans cette enceinte. Je pense au bien-être animal et à la transition écologique.

Elles se sont engagées dans les plans de filière, et je les suis au plus près. J'attends d'elles qu'elles soient au rendez-vous. L'article 13 du projet de loi prévoit d'ailleurs que le Gouvernement remette au Parlement un rapport relatif à la mise en oeuvre des plans de filière sur cette thématique précise. d'enjeux environnementaux, les filières agricoles ont un rôle majeur à jouer, de par leurs choix de production et la maîtrise de leur consommation d'intrants. La démarche agroécologique offre la réponse systémique adaptée. pour progresser de manière décisive, il nous faut cesser une bonne fois pour toutes d'opposer agriculture et environnement, reconnaître les efforts consentis jour après jour, année après année, par tous les agriculteurs, mais aussi avoir conscience de l'importance du chemin restant à parcourir et de la complexité de la transition, notamment dans un contexte où les exigences ne sont pas les mêmes dans d'autres pays. Ces difficultés ne doivent pas nous arrêter, bien au contraire. Les agriculteurs sont des chefs d'entreprise. Ils ont besoin de trouver leur équilibre économique avec les nouvelles pratiques toujours plus respectueuses des ressources naturelles, plus économes en intrants et en énergie, mais qui requièrent des changements et induisent d'autres types de coûts en termes d'investissements, de main-d'oeuvre ou de carburant. Ils ont besoin de recherche et d'innovation. Ils ont besoin de la bienveillance de leurs concitoyens et de la confiance des consommateurs. Les agriculteurs ont besoin d'un environnement porteur. Ils ont besoin d'être accompagnés et soutenus par les transformateurs et les distributeurs, les chambres d'agriculture, les collectivités territoriales, ainsi que par les financeurs, les banquiers et les assureurs. C'est toute l'approche du risque, de la rentabilité, du temps et de l'importance des biens collectifs qu'il faut revoir pour être à la hauteur de ce que la société attend de son agriculture. Au moment de passer au déploiement de tous les outils que nous avons patiemment construits depuis un an, ce dont nous avons besoin, au fond, c'est d'un retour à l'esprit des États généraux, un état d'esprit dans lequel chacun sait qu'il a sa part à prendre dans la transformation, pour qu'elle assure la pérennité de notre agriculture, sécurise notre souveraineté notre souveraineté alimentaire et soit bénéfique à tous. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire en première lecture, le projet de loi fera gagner l'agriculture si nous jouons collectif. Je regrette donc que vous ne vous associiez pas à cet élan. Hou ! La parole est

porté haut la voix de nos agriculteurs et de nos territoires. Le message avait été très bien entendu dans nos campagnes, mais il n'est manifestement pas arrivé jusqu'à la rue de Varenne, et encore moins au Palais-Bourbon

La première alerte a eu lieu en commission mixte paritaire. De mémoire de parlementaire- et j'en ai un peu ! -, c'est la première fois que j'assistais à une commission mixte paritaire échouant sur un point d'accord Alors que nous tentions de présenter des compromis sur les quelques lignes rouges restant en discussion, le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, tenu par le mandat que le Gouvernement, et peut-être même le Président refusait d'entendre la moindre de nos propositions pour centrer les débats sur un nouveau front créé de toutes pièces par la majorité : je veux bien entendu parler des modalités d'élaboration des indicateurs dans les formules de prix des contrats agricoles. Vint ensuite la nouvelle lecture, qui fut l'occasion pour l'Assemblée nationale de rétablir son texte dans sa quasi-intégralité et de balayer d'un revers de main presque tous les apports du Sénat création d'un fonds d'indemnisation des victimes professionnelles des produits phytopharmaceutiques, pérennisation du modèle coopératif, lutte contre les pratiques des centrales d'achat européennes, protection contre le chantage à la collecte, encadrement des promotions et du seuil de revente à perte directement dans la loi, pour n'en citer que quelques-uns. Plus largement, l'appel du Sénat à la retenue n'a pas été entendu. en nouvelle lecture, les députés ont réalisé le tour de force d'ajouter de nouvelles contraintes, non seulement pour les producteurs, mais aussi pour les industriels et les collectivités territoriales. Ma collègue Anne-Catherine Loisier instant. L'impression donnée peut se résumer en quelques mots : faisons la loi le plus vite possible, comme bon nous semble, comme si la sagesse du Sénat était une sorte de frein à la législation ... Permettez-moi de vous dire, monsieur le ministre,

les agriculteurs ont insisté sur la nécessité de revaloriser leur métier en augmentant leurs revenus, notamment par le renforcement de leur pouvoir de négociation contre une grande distribution trop concentrée et quelques acheteurs pas toujours bien intentionnés. Le texte prend le risque de faire l'inverse. À défaut d'accord des interprofessions et sans l'intervention de l'Observatoire de la formation des prix et des marges, les distributeurs pourront imposer aux producteurs les indicateurs qu'ils auront eux-mêmes créés, ce qui déséquilibrera encore la relation commerciale au détriment des agriculteurs. Ce texte pourrait aggraver la situation en incitant les acheteurs à fixer des prix plafonds en fonction des prix de revient qu'ils auront eux-mêmes déterminés pour les agriculteurs. Je pourrais aussi parler d'un texte menaçant l'efficacité de la médiation en introduisant la procédure du « nommer et dénoncer », qui porte atteinte à l'esprit de la coopération agricole en facilitant la sortie des associés coopérateurs au détriment du principe d'engagement, que rien n'assure que la hausse du seuil de revente à perte et l'encadrement des promotions qu'il prévoit se retrouveront bien dans le prix des produits. Il en résulte un texte auquel le Sénat ne saurait souscrire. Compte tenu de l'attitude de la majorité des députés en première lecture, aucun compromis ne sera trouvé sur les désaccords de fond restant entre nos deux chambres.

qu'il est plus que temps de répondre au désarroi de nos agriculteurs. Nous ne nous arrêterons du reste pas là, car nous créerons prochainement un groupe de suivi au sein de la commission. Très bonne idée ! C'est en effet le travail du législateur de suivre l'application des textes et d'en faire l'évaluation. La

qui alourdit dangereusement la charge des agriculteurs, mais aussi celle des industriels et des collectivités chargées de la restauration publique, aggravant les difficultés qu'il était censé corriger. L'échec de la commission mixte paritaire sur une disposition pourtant votée à l'identique dans les deux assemblées est injustifiable. nationale, au cours de laquelle les députés ont ajouté de nouveaux points de désaccord, au mépris de nos institutions, a confirmé cette volonté de refuser le dialogue, volonté préjudiciable au texte et qui trahit les engagements pris lors des États généraux de l'alimentation. Est-il besoin de rappeler que le revenu agricole, ce sont des prix, bien sûr, mais aussi des charges ? Or, non seulement la mécanique prévue au titre I n'améliorera pas le prix payé au producteur, mais le titre II ajoute de nouvelles charges. C'est particulièrement vrai en matière de produits phytopharmaceutiques. Chacun, ici et ailleurs, est convaincu de la nécessité de limiter l'usage de ces produits, à commencer par l'agriculteur lui-même : il en connaît le coût et les risques, auxquels il est le premier exposé.

Les mesures imposées, comme l'interdiction des remises, rabais et ristournes, pèseront lourdement sur les charges des agriculteurs, sans pour autant assurer une réelle réduction de l'usage des produits phytosanitaires. Ce texte fait craindre une déstabilisation d'un système vertueux de maîtrise des usages mis en place dernièrement dans le cadre des puisqu'en séparant tout conseil de la vente de produits phytosanitaires, il fait courir le risque qu'il n'y ait plus de conseil du tout. L'obligation, introduite en nouvelle lecture, de signer des chartes départementales avec les riverains pour définir des zones de non-traitement contraint, elle aussi, de façon inopportune, alors que de nombreuses démarches adaptées et fondées sur le volontariat se diffusent déjà sur tout le territoire. Ces décisions sont stigmatisantes et culpabilisantes. Elles sont en contradiction totale avec l'esprit de responsabilisation qui a prévalu lors

mesures en témoignent . L'usage des drones en terrain dangereux sera réservé à l'épandage des seuls produits autorisés en agriculture biologique ou dans le cadre d'une exploitation certifiée sur le plan environnemental, au mépris de la sécurité des autres agriculteurs, soumis aux mêmes risques. Quant à la création du fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, que le Sénat, je le rappelle, avait adoptée à l'unanimité sur proposition de Nicole Bonnefoy,

» ! Les agriculteurs ne sont pas les seuls affectés par l'inflation des contraintes introduites dans la seconde partie du texte. Les gestionnaires de services de restauration collective publique, et donc les collectivités, devront faire face, « dans le même temps », à l'obligation d'améliorer la qualité des repas servis, de proposer au moins un menu végétarien par semaine- mesure pourtant rejetée par les deux assemblées en première lecture -et de renouveler tout le matériel de cantine dès 2020, pour se conformer à l'interdiction des ustensiles en plastique les plus divers, y compris lorsqu'ils ne sont pas à usage unique, comme les boîtes ou les plateaux-repas. Je rappelle que l'objectif prioritaire affiché était de lutter contre l'usage d'ustensiles en plastique jetables ! Cette nouvelle interdiction, ajoutée au détour de la deuxième lecture, sans aucune évaluation de son impact et sans lien avec le texte, vaut pour la restauration collective, mais aussi pour tous les autres usages, qu'il s'agisse de restauration commerciale, de livraison de repas ou de distribution alimentaire et non alimentaire. Tous ces secteurs vont devoir réinvestir dans l'urgence. Les usagers paieront la facture, et que dire des industries françaises et des emplois dont l'existence est menacée à brève échéance ? Il est irresponsable de légiférer dans de telles conditions, sans étude d'impact, sans considération des conséquences concrètes, de l'explosion des coûts et des suppressions d'emplois. d'emplois. Tout laisse à penser, mes chers collègues, que la majorité gouvernementale n'acceptera pas plus, en nouvelle lecture, ce qu'elle a rejeté lors de la première, et qu'elle confirmera le durcissement du texte.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je ne reviendrai pas sur les conditions dans lesquelles s'est déroulée la CMP, dont l'échec nous conduit à siéger aujourd'hui. Les rapporteurs de la commission des affaires économiques les ont clairement exposées, et je partage pleinement leur avis et leur sentiment de gâchis

En les interdisant purement et simplement au 1 janvier 2025, ou au 1 janvier 2028 pour les collectivités de moins de 2 000 habitants, elle adopte une méthode qui me semble tant intellectuellement insuffisante que trop radicale.

Quant à l'interdiction des bouteilles d'eau plate en plastique dans la restauration collective scolaire, mon sentiment est que nous devrons réfléchir de manière beaucoup plus approfondie et globale- et moins « au coup par coup » -aux problèmes immenses que la production de ce plastique pose aujourd'hui dans le monde. Je me réjouis en revanche que l'Assemblée nationale ait conservé l'interdiction, dès 2020, des pailles et des bâtonnets mélangeurs en plastique pour boissons, que nous avions adoptée au Sénat. Je suis par contre réservé sur l'extension, à mon sens un peu trop générale, de cette interdiction aux couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers et boîtes en plastique.

Que craigniez-vous donc de la représentation nationale, monsieur le ministre, quand les associations peuvent déjà bénéficier de cette expertise de qualité ? J'en viens maintenant aux dispositions relatives aux produits phytopharmaceutiques. Sur ce sujet, notre commission avait défendu une position pragmatique, pour répondre aux inquiétudes de nos concitoyens sur les risques sanitaires et environnementaux associés à ces produits, tout en cherchant des solutions de nature à préserver l'activité des agriculteurs. Je regrette vivement que l'Assemblée nationale ait systématiquement fait le choix de rétablir les dispositions qu'elle avait adoptées en première lecture, sans aucun égard pour les améliorations objectives que nous avions apportées au texte. Je pense notamment aux articles 14, 14 et 15 traitant des pratiques commerciales relatives aux produits phytopharmaceutiques et biocides, pour lesquels notre commission avait proposé des solutions particulièrement équilibrées. À l'article 14 , l'Assemblée nationale a inséré une disposition nouvelle relative à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones habitées, qui reprend partiellement la proposition défendue par notre commission en première lecture, privilégiant une concertation préalable avant d'éventuelles restrictions administratives. Toutefois, la rédaction adoptée vise l'intégralité du territoire national, alors que notre commission proposait de mettre à disposition des acteurs de terrain un outil mobilisable selon les circonstances locales. Enfin, je regrette profondément la suppression de fait de l'article 14 A, inséré sur l'initiative de notre collègue Nicole Bonnefoy et créant un fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques.

La majorité à l'Assemblée nationale et le Gouvernement n'ont proposé, comme seule solution, que la production d'un énième rapport sur le sujet, avec un vague objectif de création d'un tel fonds à l'horizon 2020, dépourvu de toute valeur juridique. Cette décision constitue un vrai recul, monsieur le ministre, mais soyez certain que le Sénat continuera à se mobiliser pour trouver une vraie solution à ce grave problème. définitive, nous ne pouvons que déplorer le manque d'ouverture de la majorité gouvernementale sur de nombreux sujets. Nous espérions le maintien de davantage d'améliorations concrètes apportées par le Sénat, ce qui aurait permis de renforcer un texte peu ambitieux depuis l'origine. Faute de moyens et de mesures d'accompagnement suffisants, cette loi ne contribuera que de façon très modeste à la transition vers un modèle d'agriculture plus durable. La parole

après les États généraux de l'alimentation, était de rééquilibrer le partage de valeur dans les filières agricoles. Il s'agissait de répondre à une question simple : les agriculteurs pourront-ils enfin vivre décemment de leur travail ?

Aujourd'hui, nous ne pouvons que constater cet échec. Encore une fois, l'urgence que connaît le monde paysan n'est pas traitée de manière satisfaisante, et nous continuerons, au travers de débats, de missions d'information, à faire le constat d'un monde agricole qui se meurt. Car, ne nous y trompons pas, ce projet de loi sans saveur ne pose en aucun cas les bases d'un revenu paysan, alors même que cet élément apparaissait comme prioritaire à l'issue des États généraux de l'alimentation Le rétropédalage du Président de la République et du Gouvernement remet en cause une transition agricole que tout le monde semblait vouloir. Je dis bien « semblait »,

est remplacé, dans le texte que nous étudions, par le verbe « pouvoir » : nous y lisons en effet que les organisations interprofessionnelles « peuvent » élaborer ou diffuser ces indicateurs, qui « peuvent » servir d'indicateurs de référence, et qu'elles « peuvent », le cas échéant, s'appuyer sur l'observatoire. On en conviendra, entre « devoir » et « pouvoir », le champ des possibles est immense ! Alors que les paysans ont besoin d'être protégés des griffes d'un modèle économique qui les tue un peu plus chaque jour, l'État refuse de s'immiscer dans la construction des prix. Pour les syndicats- y compris la FNSEA -, « en envoyant aux acteurs économiques des injonctions à faire, l'État leur renvoie la responsabilité et refuse d'assumer son rôle de régulateur Ainsi, rien dans ce texte ne permettra la mise en place d'un prix plancher d'achat défini collectivement et prenant directement en compte les coûts de production régionaux. L'interdiction de la revente à perte et la définition d'un prix abusivement bas, ainsi que la prise en compte du revenu paysan dans la construction des indicateurs, ont été systématiquement rejetées.

ces mêmes acteurs, de l'industrie à la distribution, ne s'embarrasseront pas de scrupules dans la recherche de la maximisation de leurs profits, qu'il s'agisse de la sécurité alimentaire ou des relations commerciales, au détriment des paysans et des citoyens. sur une responsabilisation des différents acteurs est illusoire. Les agriculteurs n'y croient plus, tant la discussion interprofessionnelle est tronquée du fait du déséquilibre des forces en présence, et ce n'est pas le seul médiateur qui pourra inverser la tendance ; nous le savons toutes et tous. Nous regrettons aussi que ce texte, de manière grossière, dresse les agriculteurs contre les consommateurs, alors même que la révolution que doit connaître le monde agricole profitera à tous. à tous. Comment accepter le refus de l'étiquetage, qui renforcera la traçabilité et mettra en valeur les modes de production vertueux ? Comment accepter le refus d'inscrire dans la loi l'interdiction du glyphosate, dont on connaît la nocivité pour les agriculteurs et les consommateurs ? ? Malgré la remise en cause pure et simple du principe de précaution par le rapporteur en première lecture, nous ne pouvons minimiser la condamnation de Monsanto par la

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la nouvelle lecture de ce texte par l'Assemblée nationale a été à l'image de la CMP, où aucune discussion n'a été possible, malgré nos propositions et notre volonté de compromis au bénéfice premier des agriculteurs et des consommateurs, comme si les bonnes idées, les propositions originales, justes, pragmatiques, en phase avec les attentes de la société en matière de qualité et du monde paysan en termes de partage de la valeur, ne pouvaient émaner que du Gouvernement et de sa majorité à l'Assemblée nationale. Comme s'il fallait démontrer que la Haute Assemblée est inutile, voire gênante, elle qui représente au Parlement les territoires, sources par excellence de nos productions nourricières de base En définitive, cette conception pour le moins restrictive du dialogue aboutit à un texte plat, sans souffle, qui ne réglera rien ou presque. C'est une occasion manquée de répondre au malaise et à la déconsidération que ressentent les agriculteurs.

le texte qui nous a été soumis en nouvelle lecture, nous avons le sentiment de ne pas avoir été entendus sur l'essentiel. Nous n'avons pas été entendus sur les mécanismes de définition de la juste valeur économique qui doit être reconnue aux producteurs. Nous voulions que ces indicateurs soient validés par l'Observatoire de la formation des prix et des marges et que cet organisme public puisse en proposer lorsque les interprofessions ne le font pas. En définitive, les interprofessions agricoles seront à l'initiative de ces indicateurs, mais, en cas d'échec des négociations, il reviendra à la grande distribution et aux industriels d'en établir. Une fois de plus, ce sera le pot de terre contre le pot de fer, et rien n'aura donc changé Nous n'avons pas plus été suivis sur l'instauration du fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques- Nicole Bonnefoy y reviendra -ni sur la traçabilité des produits, exigence pourtant croissante des consommateurs.

La législation sur les relations entre coopératives et associés coopérateurs, que nous souhaitions discuter au Parlement, a été renvoyée à des ordonnances, tout comme la réforme des seuils de revente à perte. En première lecture au Sénat, 15 de nos amendements, sur 140, avaient été adoptés. La plupart d'entre eux ont été rejetés par l'Assemblée nationale. En définitive, pour le titre I, nous en restons à des aménagements de lois votées précédemment : rien de plus, rien de moins

S'agissant du titre II, les déceptions sont grandes au regard de la nécessité de prendre en compte les attentes fortes de la société. Je note comme un fait positif, malgré tout, que, contre l'avis du Gouvernement, les députés aient introduit dans le texte notre proposition de mener une étude de la définition et de la mise en oeuvre d'une prestation pour services environnementaux rendus par l'agriculture à la société. Nous en reparlerons à propos de la PAC,

Nous n'avons pas été entendus, et je vous renouvelle, monsieur le ministre, notre invitation à venir vous rendre compte de la réalité du terrain et de la dimension sociale du problème. Sur le fond, le texte qui nous est soumis aujourd'hui en nouvelle lecture reste très décevant. Il est bien en deçà du minimum que les agriculteurs étaient en droit d'attendre. Il n'améliorera pas significativement leur revenu.

L'agriculture et l'alimentation doivent être l'affaire de tous. La discussion de ce projet de loi s'annonçait, après les États généraux de l'alimentation, dans un esprit de dialogue et de conciliation. Parce qu'elle concerne plus d'un million d'agriculteurs qui animent nos campagnes, et chaque Français qui en bénéficie, la valorisation du monde agricole et de la ruralité dans son ensemble est une question vitale pour la France. Concernant ce projet de loi, les principaux objectifs fixés par le Gouvernement étaient de garantir la souveraineté alimentaire de la France et d'assurer à chacun l'accès à une alimentation saine et durable. Le texte, que nous avons longuement examiné, est le premier jalon de la mise en oeuvre de sa stratégie agricole. Tout d'abord, pour préserver la capacité de production de nos filières et garantir à la France sa souveraineté alimentaire, nous devons renverser la logique de construction des prix, favoriser le regroupement des producteurs, limiter les pratiques commerciales déloyales, telles que la revente à perte, en complément des initiatives législatives européennes. Tout au long de l'examen du texte au Sénat, le groupe Les Indépendants - République et Territoires s'est mobilisé pour défendre un modèle agricole économiquement viable pour l'ensemble des acteurs et écologiquement responsable. L'un ne va pas sans l'autre. Si l'agriculture française doit évoluer, nous devons veiller à accompagner chaque transition pour ne pas heurter une économie déjà fragile et très concurrentielle. Le titre I du projet de loi devait tout mettre en oeuvre pour permettre aux agriculteurs de vivre décemment de leurs revenus : il s'agit d'une impérieuse nécessité. À titre d'exemple, notre groupe avait proposé plusieurs orientations. Tout d'abord, nous avions défendu les enjeux propres à la filière viticole, secteur économique majeur. Nous savons qu'il est le deuxième contributeur à la balance commerciale de la France, après l'aéronautique. Malheureusement, l'Assemblée nationale a décidé de revenir sur une mesure que nous croyons pourtant juste et efficace. Le même sort a été réservé à l'amendement, adopté au Sénat de façon consensuelle, visant à lutter contre le « chantage à la collecte » du lait et le déréférencement des producteurs. Dans un deuxième temps, il s'agissait d'assurer à chacun l'accès à une alimentation de qualité, respectueuse de la santé des consommateurs et de l'environnement. Dans un climat consensuel, le Sénat avait rétabli l'objectif de 20 % de produits issus de l'agriculture biologique dans les repas de la restauration collective. Toutefois, il ne s'agit pas de sacrifier notre agriculture locale au profit d'une production certes sans pesticides, mais parcourant des milliers de kilomètres avant de parvenir dans nos assiettes. Aussi, en complément de cette mesure, avions-nous souhaité favoriser l'approvisionnement local dans la restauration scolaire, pour promouvoir l'ancrage territorial de l'alimentation. La promotion des circuits de proximité, prenant en considération le bilan carbone, est un objectif de la PAC depuis l'adoption, en juin dernier, de la proposition de résolution européenne sur l'avenir de la politique agricole commune. Il s'agit, à la fois, d'une question de souveraineté alimentaire et d'une garantie de qualité au regard des législations agricoles des pays extérieurs. L'accès à une alimentation saine nécessite une éducation suffisante du consommateur et une information lisible, fiable et accessible. Aussi ma collègue Colette Mélot a-t-elle défendu un amendement visant à rétablir à 2019 l'entrée en vigueur de l'obligation d'indication de l'origine du miel. C'était une mesure de bon sens Comme nous avons eu l'occasion de le dire en première lecture, nous pensons qu'il convient de clarifier l'étiquetage des denrées alimentaires contenant du minerai de viandes, qui représente plus de 15 % de la viande bovine commercialisée en France. Enfin, l'agriculture étant un sujet éminemment européen, nous avons défendu une disposition visant à évaluer les engagements de la France concernant les finalités de sa politique européenne et internationale en faveur de l'agriculture et de l'alimentation. Je regrette sincèrement l'échec de la commission mixte paritaire du 10 juillet dernier. Elle aurait pu permettre d'aboutir à un texte équilibré entre les deux assemblées. Nous ne pouvions pas faire l'impasse sur le dialogue s'agissant d'un projet de loi aussi important. Or la majorité des dispositions adoptées au Sénat, soutenues par l'ensemble des sensibilités politiques, ont été supprimées

Clemenceau disait que « le Sénat est la raison de la République » ; perdez la raison, et la République suivra !

l'État refuse d'assumer le rôle de régulateur de la puissance publique. Il s'agit pourtant d'une impérieuse nécessité

s'effondre, où les études sur l'impact des pesticides sur la santé s'accumulent, ce texte ne trace aucune grande orientation, aucune ligne claire pour amorcer la transition de notre agriculture vers un système vertueux, propre à rémunérer les agriculteurs et à respecter les équilibres environnementaux. Certes, il y a eu quelques avancées. On a longuement discuté dans cet hémicycle, il y a quelques mois,

je me réjouis que les députés aient voté en faveur d'une obligation d'étiquetage des huîtres permettant de distinguer les huîtres naturelles de celles nées en écloserie. C'est un combat que je soutenais depuis des années dans cet hémicycle. L'extension de l'interdiction des néonicotinoïdes est également un pas dans la bonne direction pour nos apiculteurs, dont la situation est périlleuse.

l'interdiction du glyphosate ne nous convient pas. On ne sortira pas des pesticides en se contentant d'incantations. Il en va de même du refus de définir une distance minimale par rapport aux habitations pour l'épandage de produits phytosanitaires. Tout aussi incompréhensible est le recul concernant les préparations naturelles peu préoccupantes, l'autorisation de ces solutions alternatives naturelles et sans danger continuant d'être bloquée.

d'autant que la pause estivale a apporté de nouveaux éléments, qui auraient mérité d'être discutés ici. Je pense bien sûr au procès perdu par cette société empoisonneuse qu'est Monsanto contre ce jardinier dont le cancer a été reconnu comme étant en lien avec l'utilisation du glyphosate. À défaut de débat, j'espère que le projet de loi de finances nous permettra de corriger le tir et de nous orienter enfin de manière forte et déterminée vers une nécessaire et urgente transition. Cependant, les annonces que vous avez faites hier, monsieur le ministre, sont quelque peu inquiétantes : les financements des mesures agroenvironnementales et climatiques et de la conversion vers l'agriculture biologique seraient amenés à diminuer de près de 20 %. ajoute à cela les retards de paiement des aides environnementales, l'annonce d'une baisse du budget de l'Agence Bio et la fin du financement des aides au maintien, on pourrait presque croire à une volonté de porter un coup d'arrêt au mouvement vers l'agriculture de demain, pourtant soutenu par de plus en plus d'agriculteurs et de consommateurs. Enfin, monsieur le ministre, où en êtes-vous de la mise en place des paiements pour services environnementaux, tant attendus ? La parole

Rauscent. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous commençons cette nouvelle session parlementaire en abordant un sujet qui m'est cher : l'agriculture et l'avenir de nos agriculteurs. Nous devons penser une nouvelle France agricole si nous ne voulons pas que les agriculteurs disparaissent et si nous souhaitons leur permettre de viser des marchés d'excellence en France et à l'export. Une transformation est nécessaire, car le modèle dans lequel nous sommes aujourd'hui enfermés n'est plus soutenable : le solde extérieur de l'agriculture reste certes positif, mais il est passé de 12 milliards d'euros à 8 milliards d'euros, et les Français doutent de leur alimentation. Mon groupe l'a rappelé tout au long de nos débats, le projet de loi que nous pourrions examiner aujourd'hui propose cette réforme ambitieuse dont l'agriculture française Depuis le début des États généraux de l'alimentation, l'année dernière, nous affirmons des objectifs clairs, qu'il nous incombe de graver dans le marbre : d'abord, faire en sorte que chaque agriculteur puisse vivre dignement et sereinement du fruit de son travail ensuite, rétablir la confiance entre l'ensemble des membres des filières et des interprofessions, afin de sortir des postures et d'aller vers de véritables négociations et compromis ; enfin, répondre aux nouvelles attentes des consommateurs, qu'elles soient sanitaires ou environnementales. La version du texte adoptée au Sénat nous éloigne de la concrétisation de ces objectifs. Certains articles essentiels ont été supprimés. Toutefois, au regard du bon déroulé des débats au sein de notre hémicycle et de l'ouverture d'esprit dont avait fait preuve le ministre de l'agriculture,

le titre I, j'entends les critiques de certains, qui estiment qu'il faudrait aller dans le sens d'une économie administrée, où l'État se substituerait au marché pour fixer les prix. Ce que nous proposons, au contraire, c'est que les interprofessions se coordonnent, s'organisent et se responsabilisent pour établir un partage plus juste de la valeur. Nous croyons profondément que ce sont les filières qui sont le mieux à même de construire les outils économiques adaptés à leur activité. Sans consensus au sein des interprofessions, nous n'arriverons jamais à renverser le rapport de force entre les producteurs et la grande distribution. Nous souhaitons donner aux interprofessions le pouvoir de choisir leurs indicateurs et ainsi mettre en place un cadre afin de rendre le marché plus efficace et plus juste pour les producteurs. Ce n'est pas à l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires de le faire. L'État ne peut pas imposer d'indicateurs dans le cadre d'une relation contractuelle entre deux entreprises privées. C'est cette responsabilisation des acteurs qui guide notre philosophie de l'action publique et politique. Nous avons des positions profondément divergentes sur le sujet,

assortie d'un pacte pour la préservation de l'environnement et pour le respect du bien-être animal. Si nous nous félicitons de l'accord sur l'introduction de 20 % de produits biologiques dans la restauration collective, nous regrettons vivement la suppression par le Sénat de l'une des mesures phares pour permettre une véritable refonte environnementale de notre modèle agricole veux parler de l'interdiction des remises, rabais et ristournes et de la séparation capitalistique du conseil et de la vente des produits phytosanitaires. Oui, nous pourrions refaire le débat sur le glyphosate ce serait la septième fois depuis le début de l'examen du texte. Nous sommes tous d'accord ici pour affirmer qu'il faut en finir avec cette substance. Inscrire son interdiction dans la loi servirait-il à quelque chose ? J'en doute. Le Président de la République a été très clair avec ses homologues européens : la France sortira du glyphosate d'ici à trois ans. C'est encore une fois en nous appuyant sur notre philosophie de responsabilisation des acteurs que nous souhaitons y arriver. Cette méthode trouve sa traduction concrète dans le plan de sortie du glyphosate que vous avez proposé en juin dernier, monsieur le ministre, conjointement avec l'ancien ministre de l'environnement, Nicolas Hulot.

Nous ne nous sommes pas laissé enfermer dans des débats enflammés qui n'auraient pas fait avancer les choses ; nous sommes restés paisibles et constructifs, ce qui a favorisé la qualité des débats. Nous pouvons nous en féliciter. C'est confiant en cette sagesse et à la lumière de nos débats que le groupe La République En Marche s'était abstenu en juillet dernier, dans l'espoir que les deux chambres trouvent un accord en commission mixte paritaire. Aujourd'hui, la majorité sénatoriale refuse un nouveau débat sur le texte et s'enferme dans une posture à l'égard de l'Assemblée nationale. Pourtant, près de 40 articles sur 110 ont été adoptés conformes durant la navette parlementaire.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons aujourd'hui en nouvelle lecture est décevant à plus d'un titre. Il est décevant sur le fond, car ce texte devait être l'expression des conclusions des États généraux de l'alimentation. Ce long moment d'échanges a été apprécié par tous ses participants. Leurs conclusions étaient ambitieuses et avaient suscité de l'envie et de l'espoir, non seulement pour les citoyens, mais aussi pour les agriculteurs. Comme trop souvent avec ce gouvernement, monsieur le ministre, les discours sont volontaristes et rassurants, mais les textes qui suivent sont minimalistes, voire contradictoires avec la politique annoncée. Vous allez même jusqu'à détricoter ce qui fonctionne, par exemple la sécurisation des pratiques contractuelles et des engagements pluriannuels adaptés à la filière viticole. décevant aussi sur la forme, en particulier au regard des échanges avec l'Assemblée nationale. En première lecture, les rapporteurs et les sénateurs de tous les groupes ont apporté leur contribution, en tenant compte du fait que les compromis sont essentiels au bicamérisme.

notre regard était constructif et bienveillant, le texte issu de nos débats a été totalement ignoré. Pourquoi continuer à chercher à améliorer le texte, si nos efforts décevant, voire alarmant, pour notre économie. Je suis inquiète, et mon groupe avec moi, pour nos agriculteurs et pour notre industrie. Je le disais au début de mon propos : vos actes sont trop souvent en contradiction avec vos discours.

Les députés se sont éloignés de ces objectifs. Ils ont ainsi refusé aux agriculteurs le droit de s'appuyer sur des indicateurs incontestables pour la construction de leur prix grâce à l'intervention de l'Observatoire de la formation des prix et des marges en cas de défaut de l'interprofession : c'est une erreur.

Ce contrat, associant plus d'une trentaine d'organisations agricoles et d'organismes de recherche, intègre toutes les productions, tous les territoires et toutes les filières. Il vise à développer l'innovation, le conseil, la formation et l'adoption des alternatives pour la protection des cultures afin de répondre concrètement aux attentes sociétales en matière d'utilisation des produits phytosanitaires, tout en garantissant la compétitivité de la ferme France. de ce contrat, plus de 250 solutions d'avenir ont d'ores et déjà été identifiées en matière de pratiques agronomiques, de recours au numérique, d'innovation variétale ou encore de techniques de pulvérisation et de mécanisation.

l'idée de former dans les écoles supérieures de ce territoire les élites de la Nation a été avancée. Cela leur permettrait de mieux connaître les spécificités et les enjeux du monde agricole. Je vous assure qu'elles ne seraient pas déçues ! Les agriculteurs et les techniciens seraient ravis de travailler avec elles sur les perspectives de la ferme France pour les dix prochaines années.

Je souhaite exprimer ici les regrets du groupe Union Centriste quant à la méthode adoptée par les députés de la majorité et le Gouvernement. Au Sénat, Au Sénat, les deux rapporteurs au fond, le rapporteur pour avis et l'ensemble des groupes ont travaillé sérieusement en première lecture : qu'ils en soient

Tout d'abord, nous avions souhaité donner un rôle important à l'Observatoire des prix et des marges dans la construction des indicateurs de prix. C'était une garantie de professionnalisme et d'indépendance dans cette démarche si importante pour le revenu des agriculteurs et si cruciale dans les relations entre les producteurs et les distributeurs. Au lieu de cela, les indicateurs de prix seront élaborés et diffusés par les interprofessions, et l'observatoire n'interviendra qu'Un autre

nationale d'interdire sans discernement et dans la précipitation nombre d'objets en plastique, sans même en mesurer les conséquences pour l'emploi, les collectivités, notre industrie, désaccord. Sur d'autres points encore, les députés ont eu des intentions contradictoires, et en discuter avec le Sénat les aurait sans doute aidés à retrouver le chemin de la cohérence et de la mesure.

Comment comprendre, enfin, que l'on affirme vouloir simplifier les normes tout en en créant de nouvelles encore plus contraignantes ? Manifestement, les positions de l'Assemblée nationale sont fragiles et changeantes. Les discussions sur ce texte ne sont plus possibles aujourd'hui. à quoi bon débattre de nouveau de tous les articles de ce projet de loi ? À quoi bon adopter des amendements que les députés ne liront peut-être pas ? Cette situation est plus que regrettable pour nos institutions. Le bicamérisme est le garant de la bonne construction de la loi. Pour qu'il puisse jouer son rôle, il faut un respect mutuel entre les deux chambres. C'est dans l'intérêt des Français. Ainsi, à opposer la question préalable n'est pas renoncer à nos positions ; ce n'est pas non plus abandonner nos prérogatives : c'est surtout tirer une sonnette d'alarme pour nos institutions.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Brexit, la diminution annoncée des dotations de la PAC, les conséquences possibles de l'application du CETA ou du Mercosur soumettent notre agriculture à rude épreuve. Aussi est-il urgent de lui donner les moyens d'affronter ces défis. Les États généraux de l'alimentation ont suscité beaucoup d'espoirs chez les agriculteurs, qui s'étaient vu promettre un rééquilibrage des relations commerciales et, au fond, la perspective d'une amélioration de leur revenu. En première lecture, le Sénat a recherché le compromis et l'équilibre sur bien des points. Comme nos collègues rapporteurs l'ont rappelé, la commission mixte paritaire a voulu revenir, de manière totalement inédite, sur des dispositions votées conformes dans les deux chambres je pense bien sûr à l'article 1, mesure phare de ce texte sur laquelle elles étaient parvenues à s'accorder. En effet, s'agissant de la construction des prix, l'Assemblée nationale a opéré un net retour en arrière,

la détermination d'indicateurs neutres, objectifs et indiscutables. Sans une rédaction plus contraignante, le juste retour de la valeur vers les agriculteurs risque d'être difficile resteront à la merci de la grande distribution, toujours trop concentrée. Monsieur le ministre, vous risquez de susciter une grande déception au sein du monde agricole, qui attendait beaucoup de ce texte. Les agriculteurs seront d'autant plus déçus que l'objectif initial de leur garantir un revenu décent est noyé dans un amas d'articles additionnels dont certains vont créer de nouvelles charges, normes et contraintes, irréalistes et souvent sources de déficit de compétitivité. Par exemple, s'il est souhaitable d'encourager le développement de la filière bio,

la nouvelle PAC, qui devra être porteuse d'une véritable ambition pour l'agriculture européenne et sa stratégie alimentaire. Espérons que, sur ces sujets, l'horizon sera plus clément pour nos agriculteurs, qui ne demandent qu'à vivre de leur métier, rien de plus ... La parole est à Mme Nicole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous parlons ici d'économie agricole, mais nous parlons avant tout de vies humaines, d'histoires humaines, et, à cet instant, j'ai une pensée émue et reconnaissante pour Paul François, céréalier charentais de 54 ans, président de l'association Phyto-Victimes,

Paul François vient en outre d'être durement frappé par un drame familial. Je veux ici rendre hommage à toutes les femmes d'agriculteurs qui, en silence, soutiennent leur mari ou leur compagnon, et qui, très souvent, permettent la libération de la parole de leur conjoint malade. J'ai aussi une pensée pour Fabian Tomasi, ouvrier agricole argentin de 53 ans, chargé de remplir de glyphosate les réservoirs des avions d'épandage et décédé il y a quelques jours des suites d'une neuropathie toxique sévère Fabian, que j'avais eu au téléphone, ici au Sénat, le 1 février dernier, alors que nous venions d'adopter la proposition de loi portant création d'un fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques ; Fabian qui me disait alors Remerciez le Sénat français pour ce qu'il a fait, je suis heureux. Moi, je vais mourir bientôt, mais je pense à tous les autres malades victimes qui pourront en bénéficier. J'ai une pensée pour Dewayne Johnson, jardinier municipal américain de 46 ans, atteint d'un cancer incurable du système lymphatique en phase terminale après avoir vaporisé quotidiennement des centaines de litres de Roundup et de Ranger Pro, deux poisons fabriqués par Monsanto, et qui a obtenu en première instance la condamnation de cette firme à lui payer 290 millions de dollars de dommages et intérêts. J'ai une pensée pour les salariés de Triskalia, coopérative agricole bretonne, qui se battent depuis une dizaine d'années pour obtenir la reconnaissance de leur maladie professionnelle, puis la réparation de leur préjudice, et dont l'histoire avait bouleversé tous les membres de la mission d'information sénatoriale en 2012. J'ai une pensée pour Dominique Marchal, agriculteur de 60 ans, qui souffre d'un cancer du sang et qui fut le premier exploitant agricole à obtenir la reconnaissance de son cancer en tant que maladie professionnelle. J'ai, enfin, une pensée très forte pour les familles de Yannick Chesnais, de Frédéric Ferrand, d'Alain Terrade et de Stéphane Sardin, que j'ai personnellement connus et qui sont tous les quatre décédés, victimes des pesticides, dans des souffrances atroces. Mes chers collègues, ces histoires humaines témoignent du combat que mènent seuls ces hommes et ces femmes pour obtenir reconnaissance et réparation. Leur douleur et celle de leurs familles nous obligent ; ils ne peuvent plus attendre. Monsieur le ministre,

J'ai en tête les propos d'Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé, qui avait repris en ces lieux, en janvier dernier, sans la moindre gêne, les argumentaires et les éléments de langage des firmes, en défendant des théories qui confinent au négationnisme scientifique.

Pourtant, c'était possible, car tout était prêt ! Le travail parlementaire avait été réalisé en amont depuis plusieurs années, et corroboré en janvier dernier par un rapport conjoint de l'Inspection générale

Pardonnez-moi, monsieur le ministre, mais on voit bien que tout cela n'a pas de sens, ou plutôt que tout ce qui ne vient pas d'un élu de La République En Marche est rejeté sans aucune bienveillance

En ce qui nous concerne, monsieur le ministre, sachez bien que nous interviendrons inlassablement jusqu'à la création effective du fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques que nous appelons de nos voeux. Pour toutes ces raisons, nous voterons la motion tendant à voter la question préalable. La question préalable. La discussion générale est close. Nous passons à la discussion de la motion tendant à opposer la question préalable.

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la commission des affaires économiques a décidé, lors de sa réunion du 19 septembre dernier, sur proposition de ses deux rapporteurs, de déposer une motion tendant à opposer la question préalable à ce projet de loi.

Je regrette cet état de fait, car le dialogue est toujours riche, cher Joël Labbé, et la confrontation des convictions source d'amélioration des textes- nous l'avons d'ailleurs démontré à propos du projet de loi ÉLAN. Mais dialoguer avec une assemblée sourde n'est d'aucune efficacité. Nous ne souhaitions pas allonger le processus législatif, ce qui aurait conduit à une troisième lecture à l'Assemblée et aurait ainsi retardé l'adoption de dispositions auxquelles nous croyons certes peu, mais qui seront inscrites dans votre loi et qui sont censées être utiles en vue des négociations de cette fin d'année. Je vous dois la vérité, monsieur le ministre, et pardonnez-moi d'être directe : le mépris avec lequel le texte du Sénat a été caricaturé, opposant l'« ancien monde », qui serait englué dans un obscurantisme coupable et vendu aux lobbys, au « nouveau monde », pétri de modernisme, de bonne conscience et de savoir, a été très variablement apprécié au sein de notre hémicycle, y compris par les plus modérés d'entre nous.

monde en vous ... Tous les sénateurs partagent les objectifs assignés à ce texte : augmenter le revenu des agriculteurs et améliorer la qualité de l'alimentation. En première lecture puis en commission mixte paritaire, nos rapporteurs auront auront tenté de remédier aux angles morts du texte tout en en préservant les grandes lignes, certes sans enthousiasme débordant ni adhésion aveugle, mais avec une volonté d'ouverture et de compromis qui aurait dû nous permettre d'aboutir.

Permettez-moi de rappeler qu'une commission mixte paritaire n'est pas censée créer des désaccords ; elle a au contraire pour vocation d'en résoudre. Le Sénat avait joué le jeu, ses rapporteurs proposant de nombreuses rédactions de compromis, qui n'ont même pas pu être présentées ... L'Assemblée nationale a ensuite rétabli en nouvelle lecture la quasi-intégralité de son texte, sans tenir compte des apports essentiels du Sénat. Notre assemblée avait pourtant rééquilibré ce texte sans remettre en cause sa philosophie générale, au terme d'un débat de fond de grande qualité. Je salue l'ensemble de nos collègues qui, sur toutes les travées de cet hémicycle, ont pris part à cette discussion passionnante. Une lecture attentive du nouveau texte de l'Assemblée nationale révèle même l'ajout de mesures complémentaires substantielles.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, dans ces conditions, vous comprendrez que nous ne souhaitions pas engager une nouvelle lecture de ce projet de loi : la position du Sénat a été largement détaillée en première lecture ; ce n'est pas celle de la majorité, et nous ne sommes pas en mesure de faire évoluer le texte. Comme l'ont précisé les rapporteurs, la commission des affaires économiques ne baisse pas la garde pour autant. Elle sera extrêmement attentive à la constitutionnalité du texte, à son application

prenant acte que le Sénat s'oppose au projet de loi et qu'il n'y a plus lieu d'en poursuivre la discussion, la commission

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, je ne vous le cacherai pas, je regrette de devoir discuter de cette motion tendant à opposer la question préalable. Sans revenir sur ce que j'ai dit précédemment, j'aimerais rappeler quelques chiffres. Lors de son dépôt, le projet de loi ÉGALIM comportait dix-sept articles,

Il faut y ajouter une quinzaine d'articles introduits par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture. Ce sont donc près de quarante articles qui ont été adoptés conformes pendant la navette parlementaire. Chers collègues, je ne siège parmi vous que depuis un an, mais je trouve ce ratio plutôt encourageant, et je ne qualifierai pas nos travaux d'« inutiles Le dialogue entre nos deux assemblées a bien eu lieu, on ne peut pas le nier. Malgré ces éléments chiffrés, vous vous apprêtez à adopter une motion tendant à opposer la question préalable, et ainsi à rejeter le texte sans l'examiner en nouvelle lecture. Si ce n'est là un mépris du bicamérisme, c'est à tout le moins un refus du dialogue et du principe de la navette parlementaire ; c'est comme si le travail effectué en première lecture au Sénat n'avait pas eu lieu, comme si nos équipes avaient travaillé pour rien. Pourtant, regardons ce qu'il s'est passé en juin dernier ; lorsque la discussion a lieu, nous pouvons arriver à un accord et à un consensus. Je pense à la réforme des coopératives par voie d'ordonnance davantage encadrée, à la possibilité de saisir le juge en référé en cas d'échec de la médiation,

Sur d'autres sujets- les indicateurs de prix, la réforme des coopératives, la séparation capitalistique du conseil et de la vente concernant les produits

Pour moi, choisir de ne pas examiner ce texte, c'est nier notre rôle dans la procédure parlementaire ; c'est nier notre travail d'analyse et d'approfondissement

mais on ne peut pas dénigrer ainsi le débat parlementaire et s'en exonérer. Certes, l'Assemblée nationale a retoqué un certain nombre de dispositions introduites par le Sénat vous considérez que le désaccord est si profond qu'il vaut mieux ne pas s'y pencher de nouveau. Je dois vous le dire, mes chers collègues : j'ai plutôt l'impression que la Haute Assemblée a fait le choix de couper court à toute discussion et décidé de s'enfermer dans une posture déraisonnable de refus du dialogue à coups de communiqués de presse.

ÉGALIM, CMP du projet de loi ÉLAN et projet de réforme constitutionnelle ? Est-ce à notre avantage de refuser la discussion ? Vous parlez de stigmatisation du Sénat, mais n'êtes-vous pas en train de stigmatiser l'Assemblée nationale et sa majorité élue il y a à peine un an ?

du virage environnemental que nous souhaitons prendre et de notre rapport aux animaux, vous préférez parler de la forme et utiliser ce débat à des fins purement politiciennes.

Les lignes rouges étaient connues dès l'origine. Les franchir peut rendre difficile un travail commun, mais ne remet pas en cause le bicamérisme. Parlez d'agriculture ! Ce n'est pas parce que les idées du Sénat n'ont pas été retenues que l'on peut dire que le Gouvernement et l'Assemblée nationale sont illégitimes. Le bicamérisme doit rester l'art de la controverse, et non celui du consensus mou. Le Sénat va-t-il s'enfermer dans une posture de rejet systématique des textes pour « peser » dans les débats à venir ? Permettez-moi de croire que cela n'est pas une bonne stratégie

Nous serons à l'heure pour les négociations commerciales. Nous l'avons toujours dit : nous souhaitons que les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, bref tous les acteurs des interprofessions et des filières, puissent se saisir des outils à leur disposition pour créer

j'ai participé avec un enthousiasme sincère. Rassembler autour d'une même table tous les maillons de la filière agricole pour cerner les enjeux, poser un diagnostic et élaborer ensemble les solutions : c'est comme cela que je conçois l'élaboration de la loi. Les objectifs affichés m'ont donc séduit, car je suis profondément attaché à la coconstruction et à la démocratie participative, mais les états généraux se sont arrêtés en cours de route aux portes du Sénat. La loi n'a pas été coconstruite, puisque le Gouvernement n'a tenu compte que de quelques-unes de nos préconisations, revenant au vieux clivage pourtant condamné une parodie de concertation. Nous ne nous attendions pas à voir tout point de vue divergent écarté par le Gouvernement. paritaire a échoué, car la volonté de ne pas avancer sur les propositions faites était évidente. Nous aurions aimé qu'une ligne claire se dégage dans la loi définitivement adoptée. Sinon, à quoi bon légiférer ou susciter des espoirs ? Cela ne fait qu'accentuer la défiance des citoyens envers leurs gouvernants.

celui de nos collaborateurs, mais aussi de la lassitude, à force de travailler pour rien, d'être méprisés, alors que de l'intelligence commune naît la meilleure des adhésions, à savoir l'acceptation des réformes.

Résultat : vendredi dernier, dans mon département, l'Hérault, des pomiculteurs ont tronçonné deux hectares de pommiers pour crier leur désarroi. Des centaines d'emplois saisonniers locaux vont disparaître. En effet, outre les arboriculteurs, les maraîchers et les viticulteurs sont également fortement touchés.

Le Sénat avait réalisé un travail tout à fait remarquable sur ce texte en première lecture. Je pense, comme la majorité de mes collègues du groupe du RDSE, au nom duquel j'interviens, que nous devions remettre ce texte à l'endroit et sur ses deux pieds, pour qu'il soit en cohérence avec la philosophie et les espoirs exprimés lors des États généraux de l'alimentation.

qui avaient pourtant été adoptés en des termes identiques par les deux assemblées. Je prendrai un exemple de débat que nous aurions dû avoir, qu'il nous faut avoir, car cette question ne peut se régler en catimini, par l'introduction d'une disposition boiteuse. Je vise ici les alinéas 8 à 10 de l'article 14 relatifs aux zones de non-traitement. En clair, il s'agit de jouer le sort de l'agriculture et de la viticulture et l'avenir de milliers d'emplois à la roulette russe, en invitant autour de la table des associations parfois outrancières et jusqu'au-boutistes pour réfléchir à un règlement départemental de traitement, qui s'opposera aux exploitations et qui sera à géométrie variable d'un département à l'autre. Pourtant,

Au travers de cette disposition, c'est la direction d'évaluation des produits réglementés de l'ANSES que vous discréditez. Si vous avez le moindre doute, interdisez purement et simplement la commercialisation et l'utilisation des produits ! Il faut cesser de faire planer la peur

Nous sommes surpris et navrés que le débat démocratique aboutisse à une telle impasse. Pourtant, avec les États généraux de l'alimentation, le Gouvernement avait placé haut la barre de nos espérances démocratiques. Cette grande consultation avait rencontré un vif succès et abouti à un riche vade-mecumde propositions ambitieuses. Malheureusement, dès le conseil des ministres, le projet de loi décevait ces espoirs. Malgré les tentatives de certains députés de la majorité, la première version adoptée par l'Assemblée nationale n'était guère plus à la hauteur des enjeux. Lors de l'examen du texte par le Sénat, nous avions trouvé un large compromis pour améliorer les mécanismes du titre I, notamment pour lutter contre le « chantage à la collecte » ou définir un seuil de revente à perte. Le Gouvernement, marquant une nouvelle fois le peu de cas qu'il fait du travail parlementaire, n'a pas cherché à construire sur ce compromis. Ce refus nous conduit à cette impasse démocratique et pourrait nous inciter à voter en faveur de l'adoption

Sortir en trois ans de l'utilisation de ce poison, ce n'était pourtant pas une proposition déraisonnable. Incompréhensible posture de la majorité, qui refuse d'entendre les aspirations de la société ! Plutôt que Monsanto, nous voulons des coquelicots la question préalable est aussi le moyen, pour la majorité sénatoriale, de ne pas rouvrir un débat qu'elle n'assume pas et qui la gêne. Le Gouvernement ne soulèvera pas d'objection sur ce point. Pour dénoncer le mépris démocratique du Gouvernement, sans pour autant donner à la majorité sénatoriale la possibilité de se défausser de sa responsabilité, nous nous abstiendrons. La

Ayant participé à la commission mixte paritaire, j'ai vu à l'oeuvre la tactique qui consiste à tout refuser, à ne rien écouter, à rester complètement dogmatique,

Je mets aux voix la motion n° 1, tendant à opposer la question préalable. Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi.

Le scrutin est ouvert.

lorsque nous aurons reçu le décret de M. le Président de la République portant clôture de la session extraordinaire du Parlement. Cette information sera publiée au et sur le site internet de notre assemblée.

Merci